ceux qui peinent aujourd'hui à tirer un revenu décent de leur activité et pour lesquels l'idée d'épargner n'est pas du tout d'actualité. Par ailleurs, comme cela a été dit lors de l'examen de l'article 5, il faudrait toujours garder en tête le coût de ces allégements fiscaux pour les finances publiques. Les sénateurs socialistes souhaitent toutefois rappeler qu'ils sont favorables au maintien du dispositif actuel de déduction pour épargne de précaution. Cet outil peut être intéressant pour faire face à la volatilité des revenus et à la multiplication des aléas. En revanche, en l'absence d'étude d'impact sérieuse, nous démontons l'argument selon lequel son augmentation, dans les proportions envisagées à l'article 6, viendrait répondre à une réelle demande du monde agricole dans sa diversité. Nous considérons que les éléments ne sont pas réunis pour que nous votions cet article. La parole est à M.

L'augmentation de l'ensemble des plafonds applicables à la déduction pour épargne de précaution ne pourra profiter qu'aux exploitants ayant la capacité d'épargner fortement. En effet, ce système bénéficie seulement à un nombre très réduit d'exploitations. Il semble davantage être un outil d'optimisation fiscale et sociale que de gestion des aléas. comme l'a précisé la commission des finances du Sénat dans son rapport général sur le projet de loi de finances pour 2020, seules les exploitations agricoles les plus profitables, avec les plus hauts revenus, bénéficient de la mesure. que « la situation rarement ou médiocrement bénéficiaire d'une proportion élevée d'exploitations agricoles exclura une grande majorité des exploitations du bénéfice de la nouvelle disposition ». La hausse des plafonds de l'épargne de précaution n'est pas la solution qui permettra d'encourager la compétitivité de l'agriculture française. L'effort devrait au contraire être à destination des agriculteurs qui peinent aujourd'hui à tirer un revenu décent de leur activité. De plus, le mécanisme de l'épargne de précaution permet de réduire le bénéfice agricole imposable de l'année, et donc de diminuer le montant de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales dues

toutes les auditions ont souligné à quel point elle est un outil essentiel dans la gestion pluriannuelle des aléas climatiques. Elle vient en complément des dispositifs d'assurance récolte qui ont été mis en place l'année dernière. Les agriculteurs ne s'y trompent pas, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à se saisir de ce dispositif. Selon les chiffres communiqués par l'une des banques

à une forte demande de la profession agricole, issue particulièrement des filières animales. Elles subissent de plein fouet les fluctuations du cours des céréales, qu'elles ne parviennent que très imparfaitement

En effet, la mesure viendrait baisser le coût du contrat pour les producteurs, créant une distorsion de concurrence, qu'il paraît difficile de justifier. Deuxièmement, la mesure proposée s'articule mal avec le renforcement des règles en matière contractuelle, inscrit dans le cadre de la loi Égalim, où est établi le principe du caractère pluriannuel des engagements contractuels.

Avant d'aborder les questions techniques que soulèvent ces articles, il me semble tout de même nécessaire de rétablir quelques vérités au regard du discours tenu sur les pesticides selon lequel nous serions l'un des pays les plus exigeants, et l'un de ceux qui surtransposeraient le plus ... Face à ce discours, je rappellerai simplement que l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), qui appelé l'ensemble des États membres à réduire leur consommation de pesticides, a indiqué que les plus fortes augmentations de vente de substances actives ont été enregistrées en Allemagne et en France entre 2011 et 2020. D'après l', la France serait même le troisième pays de l'Union européenne à autoriser le plus de substances actives, pour un total de près de 291 substances autorisées. Je tiens également à rappeler que 34 % de l'eau distribuée en France serait non conforme aux réglementations, notamment à cause d'une contamination par les métabolites du chlorothalonil,

vous le voyez, les exemples ne manquent pas pour prouver la quantité de pesticides dans les méthodes de production et le poids de ce lobby industriel dans de nombreuses décisions des pouvoirs publics ! Cet article 8, qui revient sur une disposition qui avait fait consensus lors de l'examen de la loi Égalim, le prouve également. Nous nous y opposerons donc avec conviction. La parole

qui autorise l'usage d'aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques. J'avais à coeur d'intervenir sur ce sujet qui touche directement mon département, où le vignoble est caractérisé, par endroits, par de fortes pentes. Le recours à des drones représente sur ces parcelles la meilleure des solutions pour la santé des opérateurs, d'une part, pour le respect et la protection de l'environnement, d'autre part. En effet, le traitement par voie terrestre est particulièrement dangereux pour les opérateurs qui en qui en sont chargés. Rappelons que procéder par voie terrestre les oblige à être directement au contact des produits et les expose à un fort risque d'accident, tant il n'est pas rare que, dans le contexte de forte pente, les chenillards

permettent des interventions efficientes et ciblées, dans le respect de l'environnement. C'est ce que confirme l'expérimentation qui s'est achevée en octobre 2022 à Guebwiller, en Alsace. Or, à l'issue de cette expérimentation, et en dépit des conclusions positives de l'évaluation réalisée par l'Anses, les exploitants concernés sont aujourd'hui sans solution. Il convient d'être vigilant et d'anticiper la fin de l'expérimentation pour les producteurs. Aussi, je suis particulièrement favorable à cet article, dont je salue la modification de bon sens rapporteure en commission en vue d'en assurer la conformité avec le droit européen. Ce sujet illustre parfaitement la manière dont l'innovation et la technologie peuvent être au service de l'agriculture, en aidant les exploitants à concilier les contraintes inhérentes à leur activité avec le respect de l'environnement. Dès lors, ne soyons pas dogmatiques et embrassons les progrès

en autorisant l'utilisation d'aéronefs télépilotés et contrôlés. Cette dérogation générale reviendrait ainsi sur une interdiction introduite par les lois Grenelle dans le droit français conformément à une directive européenne de 2009. d'information sur les pesticides adopté par le Sénat en 2012, je relevais, avec Sophie Primas, que cette technique présentait le risque d'exposer aux produits épandus des espaces situés à proximité de la zone d'épandage. La dérive, lors des épandages aériens, est d'autant plus importante que le vent est fort. Cette volatilité est un réel problème, souligné, d'ailleurs, par le rapport d'expertise de l'Anses publié à l'automne : selon ce dernier, « les applications par drone s'avèrent dans l'ensemble moins efficaces que celles par pulvérisateurs classiques ». Par ailleurs, le même rapport constate que « les niveaux de contamination des mannequins, placés à une distance de la parcelle de 3 et 10 mètres, sont supérieurs lors d'une pulvérisation avec un drone en comparaison avec un atomiseur à dos ». Alors que cette étude renforce les inquiétudes sanitaires et remet même en question l'efficacité de cette technique, de cette technique, il n'est pas sérieux de revenir sur cette interdiction. Il y va de la protection de la santé de nos agriculteurs, qui sont les premières victimes des pesticides. Les dérogations à l'interdiction de l'épandage aérien qui existent d'ores et déjà doivent rester l'exception et répondre à des motifs très précis. Pour ces raisons, nous vous demandons de supprimer cet article, qui, s'il était adopté, remettrait en cause un acquis législatif solide pour la défense de notre environnement.

ans et que les insectes et les pollinisateurs disparaissent de manière dramatique. Nous faisons partie des pays qui, comme d'autres, peinent à maintenir la biodiversité dans leurs milieux agricoles, alors même que produire autrement est aujourd'hui une question de survie du modèle agricole lui-même. Au regard de ces éléments, du manque d'informations sur les impacts potentiels sur l'environnement et en application du principe de précaution, il nous paraît nécessaire de poursuivre les études à ce sujet et de mettre en place des procédures d'évaluation de risques sur l'environnement, en particulier sur les pollinisateurs, qui, nous le indispensables à notre système agroalimentaire. De plus, nous ne pouvons avec certitude écarter le risque sur la santé des agriculteurs et des salariés agricoles eux-mêmes. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

une potentielle dérive, dans les sédiments, 3 à 5 fois plus importante pour les pommiers. L'Anses précise que les drones entraînent un courant descendant dû à leur rotor, qui représente des risques différents des technologies préexistantes. Elle montre un dépôt de pesticides irrégulier sur les cultures, qui peut exposer les travailleurs à des quantités de produits problématiques. Comment, dans ces conditions, proposer d'ouvrir à des usages plus larges ? L'expérimentation proposée ne nous semble pas conforme à l'interdiction des épandages aériens prévue par le droit européen. Elle va à rebours d'une politique de sortie de l'usage des pesticides que nous appelons de nos voeux, cependant qu'elle expose nos

l'avis de la commission ? L'usage des drones en agriculture ne fait pas consensus, comme le prouvent ces amendements de suppression. Je vais essayer de m'en tenir aux faits et de ne pas trop verser dans l'opposition la rédaction initiale envisageait une autorisation générale de l'utilisation des drones. Notre commission a largement fait évoluer le dispositif, en le transformant en une expérimentation sur

à la fois le travail d'évaluation et le travail de recommandation sur l'utilisation des drones plaide en faveur de cette expérimentation.

que vous l'accepterez pour maintenir la riziculture et pour maintenir cet équilibre qui nous est si cher en Camargue. La parole est à M. Guillaume Gontard,

l'article concernant les travailleurs, que « plusieurs études montrent que les dépôts sur les cultures présentent une variabilité supérieure après utilisation de drones en comparaison avec les matériels d'application classiques. Ainsi, la question de l'impact de la quantité des dépôts sur les cultures sur l'exposition des travailleurs se pose ». Il faut savoir s'arrêter là et se dire que ce

Le présent amendement, déposé par notre collègue Henri Cabanel, a pour objet de préciser que les drones mentionnés à l'article 8 ne peuvent être des drones dont la motorisation est thermique. Il faut rappeler, dans un premier temps, que cet article vise à déroger au principe d'interdiction des traitements aériens pour les produits phytosanitaires dans les États membres de l'Union européenne. Si cette procédure d'exception ne s'étend qu'aux aéronefs télépilotés ou contrôlés par intelligence artificielle, pour la pulvérisation de précision de produits phytopharmaceutiques sur des terrains agricoles en pente ainsi que pour l'agriculture de précision, il me semble nécessaire de rappeler que le plus haut niveau d'exigence environnementale indispensable à l'autorisation de cette dérogation passe aussi par la limitation des émissions directes en gaz à effet de serre. En ce sens, il n'est pas concevable que la dérogation prévue par le présent article puisse autoriser le recours à des aéronefs à motorisation thermique, d'autant plus dans le contexte de la transition énergétique et écologique. Il faut rappeler que l'autonomie reste l'un des points faibles des drones et peut varier selon les conditions météorologiques ou les manoeuvres à effectuer. L'une des possibilités d'extension serait de passer sur des systèmes de motorisation

Au regard de l'interdiction des applications de produits phytopharmaceutiques par hélicoptère et des limites associées au passage des pulvérisateurs, le recours à des drones de pulvérisation est envisagé comme une alternative pouvant présenter de multiples avantages.

par le groupe socialiste. Il s'agit de limiter la réintroduction de cette expérimentation à un dispositif proche de celui qui avait été voté dans le cadre de la loi Égalim, afin que la pulvérisation par drone ne puisse être autorisée que pour les autorisés en agriculture. En effet, nous tenons à rappeler que nous souhaitons avant tout le maintien de l'interdiction générale de l'épandage aérien de pesticides, avec, comme seule exception, les cas de dangers sanitaires graves ne pouvant être maîtrisés par d'autres moyens, comme le précise actuellement l'article L. 253-8 du code rural.

à l'usage des pesticides. Il s'agit donc de ne s'affranchir ni de l'évaluation de l'Anses ni du droit européen. Toutefois, je m'interroge sur l'opportunité de laisser à l'appréciation d'une autorité administrative le soin d'ouvrir la possibilité au ministère de délivrer ou non des autorisations d'utilisation de drones pour certaines productions. Une expérimentation de cinq ans doit être menée. Il sera bien temps de légiférer de nouveau à la lumière des conclusions qu'on pourra en tirer. Je m'en remets donc, pour cet amendement, à la sagesse de notre assemblée.

au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

pour valoriser les apports environnementaux de l'agriculture en général et des agriculteurs en particulier- les reconnaître et les payer.

Les gouvernements qui se sont succédé ces derniers temps ont un peu avancé en ce sens, notamment en créant un fonds de 150 millions d'euros dans le cadre du plan biodiversité pour développer les PSE.

PSE sont un levier trop peu mobilisé pour encourager et aider financièrement les agriculteurs à mener des actions visant à maintenir ou à restaurer des services écosystémiques. J'ai également le souvenir qu'une précédente demande de rapport avait été faite un amendement adopté dans le cadre de la loi Climat et résilience, sur l'initiative de la rapporteure Anne-Catherine Loisier, et relatif à l'extension des PSE à la forêt.

dispose que la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation a pour finalité de reconnaître et mieux valoriser le stockage de carbone dans les sols agricoles. Cet

vise à ce que la politique d'aménagement rural traite la transition des exploitations agricoles de manière globale et systémique, en prenant comme fil conducteur le changement climatique. Pour assurer leur viabilité, les exploitations doivent s'inscrire dans une démarche d'atténuation du changement climatique, au travers des réductions de leurs émissions de gaz à effet de serre et de l'adaptation au changement climatique. La réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité de l'exploitation agricole et d'un plan de transformation de cette dernière, choisi par l'agriculteur, permettra aux exploitations agricoles de contribuer de manière pérenne à la lutte contre le changement climatique.

La dynamisation, la modernisation, l'attractivité et la durabilité de notre modèle agricole ne pourront être atteintes sans prendre en compte l'évolution des pratiques agricoles que le changement climatique ainsi que les transitions écologique et climatique induiront. Le besoin de visibilité et d'accompagnement est essentiel dans ce contexte soumis aux changements climatiques, sociaux ou démographiques.

prie de m'excuser ... Cet amendement vise à rappeler un élément fondamental : le fait de considérer l'impact carbone de l'agriculture sans prendre en compte la biodiversité et les autres dimensions environnementales est une erreur qui produit de nombreux effets pervers. Il semble davantage pertinent d'évaluer globalement la performance environnementale de l'exploitation agricole, plutôt que sous le seul angle de

étendre le dispositif, globalement, à la protection de la biodiversité, à la qualité de l'eau et à la qualité de l'air, et à supprimer la référence à la qualité agronomique des sols,

Il est important d'encourager la relocalisation de l'alimentation, la traçabilité et la transparence pour le consommateur. Un affichage des trois premiers ingrédients ne permettra pas d'atteindre cet objectif. Quel

établissements qui livrent à domicile, mais n'ont pas de salle pour consommer sur place. Un décret a bel et bien été pris pour rendre obligatoire l'indication de l'origine des viandes en

L'alimentation ultratransformée est en grande partie responsable de ce fléau et l'état actuel des connaissances appelle à la mise en place de premières actions préventives de santé publique. En s'appuyant sur l'usage du Nutri-score, qui ne fait plus débat aujourd'hui, des actions ambitieuses visant les produits trop gras, trop salés et trop sucrés pour lesquels des preuves de nocivité sont indubitables et communément admises doivent être mises en place. D'après l'OCDE, une réduction de 20 % de l'apport calorique des aliments riches en sucre, en sel, en calories et en graisses saturées permettrait de prévenir 582 000 cas de maladies non transmissibles d'ici à 2050 en France. Pour que le consommateur puisse facilement et rapidement faire le tri dans les rayons de supermarchés, les denrées alimentaires présentées à la vente doivent comporter un étiquetage permettant de bien l'informer, en particulier lorsque celui-ci s'apprête à consommer un aliment ultratransformé. À ce jour, ces aliments représentent dans notre pays probablement de 40 % à 50 % de l'offre actuelle en supermarché, et seraient, selon les chercheurs, la première cause indirecte de mortalité précoce dans les grandes villes, responsable en grande partie de la stagnation de l'espérance de vie en bonne santé, laquelle est inférieure à 65 ans pour les hommes et les femmes. Les ingrédients et additifs cosmétiques utilisés dans ces aliments sont en réalité des substances alimentaires non habituellement utilisées en cuisine, que les industriels utilisent pour limiter les qualités organoleptiques d'un aliment brut et de leurs préparations culinaires, ou pour masquer les défauts d'un produit. En outre, on ne sait encore que peu de choses des effets cocktail potentiellement délétères de ces additifs sur le long terme, ainsi que de leur action sur la flore microbienne. Il est donc urgent de réguler un tel commerce, mais des dispositions transitoires afin de ne pas perturber les acteurs du commerce et de la distribution,

de qualité durable. Sont concernés : l'État, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics. L'article 11 assouplit la définition des produits durables et de qualité qui doivent composer une part significative de l'offre alimentaire en restauration

ses services s'intéressent à « la composition du produit, à ses caractéristiques visuelles, olfactives et gustatives ou à certaines règles de fabrication le champ retenu est beaucoup trop large et n'offre pas les mêmes garanties de durabilité et de qualité que les produits estampillés d'un signe de qualité, d'un écolabel, d'une mention « fermier » ou « produit à la ferme », ou encore issus de l'agriculture biologique.

deux exemples. Le certificat « agneau de qualité », de la Fédération bétail de qualité Bourgogne, domiciliée en Côte d'Or- chez Anne-Catherine Loisier -, garantit que l'agneau est élevé avec sa mère pendant 60 jours, avec une alimentation complémentaire, et qu'il est élevé pendant 270 jours au maximum.

Je soutiens ces amendements. Comme le ministre l'a souligné, en Île-de-France, des plans alimentaires territoriaux sont en cours d'élaboration dans la plupart des collectivités.

Labbé. Par cet amendement, nous souhaitons répondre aux difficultés d'application de la loi, en nous dotant d'outils de dynamique territoriale. Pour affirmer une véritable volonté politique sur l'application de cet article et lever les blocages, cet amendement vise à ce que soit nommé un sous-préfet référent pour l'application de la loi dans chaque département. pourrait faire remonter les difficultés des collectivités locales et organiser la concertation entre les acteurs. Nous en sommes convaincus, il faut faire appliquer cette loi et non proposer de revenir en arrière

Ces contrôles devront être réalisés par des laboratoires habilités, et non par les services déconcentrés de l'État. Le ministre m'objectera sûrement que la révision à venir de la directive Miel de 2001 nous donnera, enfin,

Premièrement, concernant les miels issus d'assemblages, les analyses effectuées sur les produits finis ne permettent de contrôler ni l'origine géographique et florale ni l'absence d'adultération. Seules des analyses réalisées avant assemblage peuvent détecter l'intégralité des fraudes. de ces amendements introduirait une situation de concurrence déloyale concernant les miels commercialisés sur le marché français. En effet, les opérateurs français seraient contraints de réaliser les analyses que vous réclamez, alors même que leurs concurrents,

C'est un vrai sujet. Il faut aussi penser à tous les apiculteurs qui perdent à peu près 30 % de leurs abeilles tous les ans. Si d'autres agriculteurs perdaient 30 % de leur cheptel tous les ans, il est évident que cela deviendrait un sujet

Il rappelait aussi que les États membres avaient le droit de fixer des normes plus élevées que celles qui étaient définies par la directive. En ce sens, toute surtransposition n'est pas nuisible en elle-même et peut résulter d'un choix

la remise en cause de toute ambition en matière environnementale et de progrès vers une réelle agroécologie. Pire, c'est une véritable régression et le choix de la logique du moins-disant environnemental et sanitaire. Pourtant, en France, 85 000 tonnes de pesticides sont répandues chaque année. Notre pays est le premier consommateur européen et le troisième mondial.

n° 74. Cet amendement vise également à supprimer l'article 12 de cette proposition de loi, qui introduit un principe de non-surtransposition des directives européennes en l'absence de motif d'intérêt général. Tout d'abord, nous avons de réels doutes sur la rédaction de cet article.

De même, la notion d'exigence minimale pour la transposition est particulièrement inquiétante sur le fond, car elle reviendrait à contraindre le gouvernement français et le législateur à se positionner sur les critères les plus faibles. Pourtant, nous savons bien que les négociations européennes, souvent longues et complexes, aboutissent régulièrement à des échelles adaptables pour convenir à la grande majorité des États membres. Adopter un tel article reviendrait à être le moins-disant possible dans les transpositions du droit européen, qui va du sanitaire au droit du travail, et à affaiblir considérablement la position française dans les débats européens. pourtant indispensable que la France tienne une position forte pour demander une harmonisation des normes européennes à la hausse pour l'ensemble des États membres. L'harmonisation est le seul moyen pour éviter les distorsions de concurrence. L'objectif visé par cet article n'est donc pas le bon.

Il réduit l'analyse des politiques publiques aux seules conséquences financières. N'est-ce pas caricatural ? De plus, présenter les surtranspositions comme une problématique majeure de l'agriculture française, comme le fait le rapport qui est à l'origine de cette proposition de loi, n'est-ce pas une caricature ? Un rapport du Gouvernement de 2022 estime pourtant que les surtranspositions sont rares et que, quand elles existent, elles sont pleinement assumées. Encore une fois, on peut se demander de quel côté est la caricature.

des aliments (Efsa) rejoignent celles de l'Anses. N'est-ce donc pas de la caricature que de crier à la surtransposition, comme on a pu l'entendre dans le débat public ? Pour nous, et comme le rappelait ce rapport, aller plus loin ce rapport, aller plus loin que le droit européen est légal et légitime, notamment pour protéger les citoyens et notre environnement. Cet article cherche à contraindre cette possibilité ; nous estimons au contraire que la France doit être leader sur ces sujets, ce qui permettrait par ailleurs d'anticiper les problématiques à venir. très important, qui vise avant tout à tirer la sonnette d'alarme sur les surtranspositions qui affectent massivement le monde agricole

pour éviter les distorsions de concurrence ». Alerter sur les surtranspositions ne signifie pas pousser au moins-disant. Cela revient à insister sur la nécessité de prendre garde, avant d'adopter des mesures pénalisantes pour notre agriculture sans aucune concertation européenne ni évaluation des conséquences et des effets de bord. Poser un principe de non-surtransposition, comme l'ont fait d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, est un signal clair envoyé au Gouvernement. Il ne s'agit pas de priver le Parlement de son droit fondamental à légiférer ; il n'en a jamais été question et ce serait juridiquement impossible. C'est

de demander au Conseil d'État d'identifier dans ses avis les surtranspositions et de demander au Gouvernement de s'en expliquer. Cet article améliore l'information du Parlement. Les Allemands le font, je ne vois pas pourquoi nous ne le pourrions pas ! Quel

le prônent certains de mes voisins dans cet hémicycle, il est clair que nous reviendrons rapidement aux famines du Moyen Âge. Nous aurons toujours des insectes, des bactéries, des champignons prêts à dévaster nos cultures.

vote. Soyons raisonnables ! Le Président de la République a dit : « Il n'y aura pas d'interdit sans solution. » Il a raison. Il a raison. Voilà bien des années que les néonicotinoïdes sont utilisés sur la betterave, qui n'est pas une plante mellifère.

et, de l'autre, une agriculture qui ne pense qu'à ramasser du pognon, quitte à jouer avec la santé et le bien-être de nos concitoyens. Nos collègues

À l'inverse de la logique proposée à l'article 12, nous proposons ici un principe de non-« sous-transposition » et de lutte contre les sous-réglementations en matière environnementale, sanitaire et de protection sociale. interroger sur une bonne harmonisation du droit de l'Union européenne entre les États membres et sur une juste articulation entre le droit national et le droit communautaire. Or, en mettant l'accent sur les surtranspositions, cet article occulte un pan entier de la réflexion : le fait que la France est également concernée par des sous-transpositions ou des sous-réglementations.

Dans une décision du 15 novembre 2021, le Conseil d'État a enjoint au Gouvernement de prendre, dans un délai de six mois, les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'utilisation de pesticides soit effectivement restreinte, voire interdite, dans les zones classées Natura 2000 pour se conformer au droit européen. La Commission européenne a également estimé prendre très au sérieux les potentielles infractions à la directive-cadre sur l'eau liées aux projets de stockage d'eau qui se développent sur le territoire français.

Je mets aux voix l'article 19. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Nous proposons de compléter le contenu du rapport relatif à la mise en oeuvre des clauses miroirs, dont on parle si souvent, plus précisément en ce qui concerne l'article 44 de la loi Égalim. Ce dossier n'avance pas. Les moyens affectés par l'État pour protéger notre agriculture de la concurrence déloyale des produits importés qui ne sont pas conformes aux exigences que, à raison, nous nous appliquons appliquons sont bien trop faibles pour permettre à l'administration de mener à bien sa mission. L'instauration de clauses miroirs aux frontières du marché intérieur serait pourtant un moyen de protéger notre agriculture de la concurrence déloyale, cela est démontré dans le rapport d'information du Sénat sur les retraits et les rappels de produits à base de graines de sésame importées d'Inde ne respectant pas les normes minimales requises dans l'Union européenne et dans le rapport sur le projet de loi de finances pour

est l'un des éléments permettant de construire une véritable compétitivité pour notre agriculture dans ses dimensions économiques, sociales, environnementales et sanitaires. Nous proposons que soit

ou de libre-échange. Sans régulation des marchés agricoles et sans sortie de ce secteur des accords de libre-échange, la construction de la compétitivité environnementale, sociale, économique et sanitaire de notre agriculture sera nécessairement mise à mal par la concurrence de productions moins-disantes. Penser que les agriculteurs français pourront rivaliser avec leurs concurrents à l'échelle mondiale est un leurre. Une telle rivalité n'est en outre pas souhaitable, car la compression des normes et des charges se fait au détriment de la protection sociale des travailleurs et de l'environnement.

des produits phytopharmaceutiques, une balance détaillée des bénéfices et des risques sanitaires, environnementaux et économiques. En commission, la rapporteure a proposé de réécrire le dispositif, estimant que l'Anses ne pourrait pas assumer cette mission, et donné au ministre de l'agriculture le pouvoir de suspendre une décision du directeur général de l'Anses sur le fondement de cette balance bénéfices-risques. L'article 13 prévoit également d'introduire un délai de grâce systématique en cas de retrait d'une AMM pour permettre, dans un premier temps, et pendant six mois, de continuer à vendre et distribuer ce produit, puis, dans un second temps, de continuer à l'utiliser, à le stocker ou à l'éliminer pendant une année supplémentaire. Les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s'opposent fermement à ces deux propositions,

D'une part, nous estimons que l'Anses est une agence d'expertise scientifique indépendante, dont le rôle est notamment d'évaluer l'impact d'un produit sur la santé humaine et l'environnement. Il semble inenvisageable que ses décisions puissent être dictées

pose aussi de graves questions en matière de sécurité sanitaire et environnementale. Rien, dans cet article, ne va dans le bon sens. Une fois de plus, nous avons le sentiment que, derrière la recherche de compétitivité, il y a une volonté de déréguler et de déréglementer.

mais de procéder à une analyse bénéfices-risques, de vérifier si les molécules qui sont en cause sont autorisées ou pas dans d'autres pays européens, s'il existe des solutions de repli et d'évaluer les conséquences sur les filières et sur l'industrie agroalimentaire.

au coeur des débats sur cette proposition de loi. J'ai déjà fait part de mes réticences sur un certain nombre de dispositions concernant l'usage des pesticides. Comme je l'ai expliqué lors de la réunion de la commission des affaires économiques, les modifications qui ont été introduites en commission sont pour moi une ligne rouge, car elles induisent un durcissement du dispositif. La version initiale de cet article préservait la souveraineté de l'Anses, et ce malgré l'introduction d'un calcul bénéfices-risques. En offrant au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire un droit de veto sur ses futures décisions, les modifications introduites en commission retirent son pouvoir décisionnaire à l'Agence. Confier la décision finale de l'interdiction d'un produit phytosanitaire au ministre présente le risque que les arbitrages ne se fassent pas dans le but de défendre le seul intérêt général. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai fait en commission des affaires économiques, je voterai contre l'article 13. La parole est à M.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

par les politiques publiques. Nous proposons aussi de chiffrer la part des dépenses publiques qui financent ces pratiques néfastes. Une étude des financements publics liés à l'utilisation agricole des pesticides en France a été publiée en 2021 par la Fondation Nicolas Hulot et le bureau Basic : elle montre que moins de 1 % des dépenses publiques contribue réellement à la réduction de l'usage des pesticides. Ces données sont intéressantes pour orienter notre politique agricole. Nous proposons enfin de chiffrer l'ensemble des externalités positives, qu'on appelle aménités, dont nous bénéficions du fait des pratiques alternatives agroécologiques. L'agriculture biologique, notamment, protège l'eau, les sols, la qualité de l'air, la biodiversité, les pollinisateurs. Ces données

une fois que tous les leviers de sobriété ont été mis en oeuvre, notamment les pratiques agronomiques permettant de retenir l'eau dans les sols. Je rappelle que 93 % de notre agriculture est une agriculture pluviale, qui n'a donc pas besoin d'irrigation. Déclarer ces projets d'intérêt général majeur sans aucun encadrement ni garde-fou ne nous semble pas la solution. Certes, l'article a été modifié en commission pour tenter d'atténuer la mesure, en l'articulant avec le principe de l'usage partagé et les hiérarchies des usages de l'eau, mais cette précision est insuffisante. Si l'irrigation est nécessaire dans certains cas, elle doit être conditionnée à des pratiques agroécologiques et au soutien à la souveraineté alimentaire, et non être déclarée comme présumée d'intérêt général majeur. L'objectif est de placer l'usage agricole de l'eau au même niveau que l'eau potable et l'usage sanitaire, ainsi que le bon fonctionnement des milieux aquatiques déjà largement mis à mal. Des alternatives à l'actuelle généralisation de l'irrigation existent produire sur des sols vivants et avec des principes d'agroécologie. La priorité, face à la raréfaction de la ressource en eau, doit être de discuter des changements à opérer. La répartition des volumes d'eau d'irrigation entre les filières et le rôle de ces dernières au sein de stratégies territoriales doivent retenir toute notre attention. La

les sénateurs de mon groupe considèrent dans leur très grande majorité qu'il serait très difficile de traiter ce sujet au détour de cette proposition de loi, sans étude d'impact ni concertation. Sur le fond, nous regrettons le parti pris beaucoup trop marqué de cet article 15, qui propose de reconnaître dans la loi, par principe, le stockage de l'eau en agriculture comme d'intérêt général majeur. Au vu du contexte sociétal et politique extrêmement tendu sur cette question, il ne nous semble pas judicieux d'inscrire un tel principe dans la loi au détour de l'examen d'un texte qui, nous le rappelons, n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact. La question des retenues d'eau en agriculture est complexe. Seule une solution équilibrée et durable pourra apaiser les tensions et répondre aux attentes des différents acteurs concernés par ce type de décision.

pourront émerger. Dans cette attente, il nous semble totalement imprudent d'inscrire dans la loi des positions aussi définitives. Nous vous proposons donc de supprimer cet article. La parole est à M.

redevenue une problématique structurante du débat public, alors que nous nous étions habitués à une certaine abondance et à une relative facilité. L'agriculture est en première ligne, puisque

territorialisation de la politique de l'eau. Il a réaffirmé l'importance du respect de l'équilibre entre prélèvements et ressources et annoncé l'accompagnement de la création d'un fonds hydraulique

de la multiplication des actions en justice et de la capacité qu'ont certains acteurs, qui ne sont pas toujours implantés localement, d'alourdir les procédures et d'allonger les délais de mise en oeuvre. alimentent l'agribashing et estiment parfois être mieux placés pour décider des stratégies locales de gestion de l'eau que les citoyens et les élus. Quel est l'avis de la commission ? L'équilibre

qui consacre la gestion équilibrée de la ressource sans interdire le stockage. Le paragraphe 7 de l'article 4 de la directive-cadre sur l'eau de 2000 permet de déroger au principe de non-détérioration de l'état d'une masse d'eau ou de ne pas atteindre les objectifs de bon état dans le cadre

M. Daniel Salmon. Je reviens sur un point : ce texte ne propose pas de qualifier l'alimentation en eau potable ou le fonctionnement des milieux aquatiques comme étant d'intérêt général majeur. Il y a pourtant une hiérarchie dans les usages de l'eau, que tout le monde connaît.

Je mets aux voix l'article 15. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste-Solidarité et Territoires. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Merci, d'être plus longuement expertisé, puisque les ouvrages de prélèvement et de stockage de l'eau sont soumis à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux, activités (Iota). Cette nomenclature permet de savoir si un ouvrage doit faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration. L'amendement mentionne le volume de la réserve, qui est certes un critère de la nomenclature, mais d'autres éléments doivent être pris en compte tels que la superficie du plan d'eau, sa hauteur, son mode d'alimentation ou encore la zone dans laquelle la retenue est installée.

M. Daniel Salmon. Nous estimons que les mégabassines ne constituent pas un modèle efficace et durable. Nous pouvons d'ailleurs le constater, comme je le disais tout à l'heure, en Espagne, où le recours aux réserves de substitution est important et où les ouvrages peinent à se remplir

Au sens des instructions ministérielles du 7 mai 2019, les PTGE ne concernent pas uniquement les ouvrages et usages agricoles de l'eau- ce que nous inscrivons ici dans le code de l'environnement. Les modalités actuelles de concertation sur les PTGE ne permettent pas de penser de façon partagée l'usage de l'eau.

Afin de rendre les PTGE plus efficaces, nous donnons toute leur place aux mesures que sont la recherche de la sobriété des usages, les changements de pratiques agricoles et les solutions fondées sur la nature aux multiples cobénéfices

la référence à l'instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative aux PTGE. La loi n'a pas vocation à renvoyer à des instructions gouvernementales l'application d'une mesure. Par ailleurs, cet amendement est incomplet dans la mesure où l'instruction susmentionnée a d'ores et déjà été complétée par un additif

l'ensemble des acteurs entendus lors des auditions m'ont invitée à ne surtout pas rigidifier les PTGE, qui sont des outils agiles de concertation locale. Cet amendement entend dresser une longue liste des parties prenantes aux PTGE, ce qui n'est pas souhaitable. Il faut laisser à l'intelligence des territoires le soin d'organiser leurs propres concertations.

de prélèvement et de stockage d'eau. Alors que les questions relatives à la création de ces ouvrages sont source de nombreuses tensions dans les territoires, il n'apparaît pas opportun de limiter l'accès à la justice. Le Le véritable outil pour éviter l'extension des contentieux est une concertation large et sincère- nous en parlions tout à l'heure. De plus, cet article présente un risque d'asphyxie des CAA, ce qui serait contraire à l'objectif affiché de réduction de la durée des contentieux relatifs à ces

en reconnaissant que les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, les recours contre les projets d'ouvrages de prélèvement et de stockage d'eau. À l'instar de ce que nous avons dit concernant l'article 15, nous estimons qu'aucune décision ne doit être prise hâtivement sur le sujet sensible de l'eau, plus particulièrement sur la question du stockage en agriculture. De plus, une nouvelle fois, une prise de position aussi tranchée vient nécessairement faire écho à l'actualité et ne manque pas de soulever une vive opposition de la part du monde associatif et citoyen. À ce sujet, le secteur associatif est formel : il n'y a pas de prolifération des contentieux. Si certains projets sont particulièrement médiatisés- je pense évidemment à Sainte-Soline -, il ne faut pas en tirer de mauvaises conclusions ni en faire des généralités non pertinentes. Par ailleurs, nous ne partageons pas la philosophie ambiante, portée notamment par le Président de la République, considérant que tout doit être accéléré et que les outils de contrôle démocratique, de ces projets sur notre environnement, doivent être remis en cause. Ce n'est pas la conception que nous avons de l'agriculture de demain ni d'ailleurs de la gestion de l'eau en tant que bien commun. Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à l'article 17 et en demandons la suppression. La

réalisé par notre collègue Nicole Bonnefoy en 2012 et d'une proposition de loi de 2013. Revenir sur de telles interdictions va à l'encontre de l'histoire et à rebours de la volonté, affichée par les pouvoirs publics, de diminuer la consommation de pesticides en France. L'article acte un recul pour la protection des sols et de la santé des Français, alors que la transition agroécologique devrait être au coeur de nos préoccupations. S'agissant de la séparation des activités de vente et de conseil, je tiens à rappeler l'existence d'un risque de conflit d'intérêts, dès lors qu'il reviendrait aux mêmes personnes

Je tiens d'ailleurs à rappeler que, dans le cadre de la loi Égalim, les rapporteurs de l'époque, Michel Raison et Anne-Catherine Loisier, s'étaient opposés à la suppression J'espère que, par cohérence, il en ira de même aujourd'hui. En tout état de cause, il nous semble impensable de soutenir un tel article, dont nous proposons la suppression. La parole est à M.

Or ces interdictions avaient été instaurées pour réduire l'utilisation des pesticides. Le cumul des activités de vente et de conseil pour les pesticides entraîne entraîne des conflits d'intérêts et des conseils orientés pouvant conduire à une surutilisation de ces mêmes pesticides et,, à une augmentation des risques de contamination pour les pollinisateurs. Pire, vous revenez sur une disposition qui a déjà été affaiblie. Ainsi, la séparation capitalistique des structures économiques n'est pas totale, puisqu'a été introduite la possibilité que 32 parts d'une structure de conseil soient dans les mains de structures de distribution. Les structures de conseil pourront donc toujours être influencées par les vendeurs de pesticides. La parole

de 2018 qui ne sont entrées en vigueur qu'en janvier 2021. Il est nécessaire de rappeler que l'esprit de cette seconde mesure était de prévenir tout risque de conflit d'intérêts résultant de la coexistence chez un même opérateur des activités de conseil et de vente pour les produits phytopharmaceutiques et de garantir aux utilisateurs professionnels un conseil annuel individualisé,

dans les méthodes alternatives, le déploiement des nouvelles technologies ou les biocontrôles, pour soutenir les agriculteurs dans la trajectoire de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, tout en préservant leur compétitivité. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article. La parole est à M.

aujourd'hui de revenir sur cette disposition. Nous souhaitons nous opposer à ce recul majeur pour l'environnement et pour les agriculteurs. Le cumul des activités de vente et de conseil pour les pesticides entraîne des conflits d'intérêts et des conseils orientés pouvant conduire à une surutilisation des pesticides,

pour l'autonomie des exploitations, pour leur performance économique et pour nos ambitions collectives de sortie des pesticides. Alors, n'envoyons pas, en adoptant cet article, un signal de recul sur le sujet des produits phytosanitaires

bien avant la séparation du conseil et de la vente, de nombreux garde-fous avaient été mis en place. Ainsi, les vendeurs comme les conseillers devaient détenir un agrément spécifique délivré par l'autorité administrative, en plus du certificat

insinuant que les agriculteurs utiliseraient à dessein plus que ce qui est nécessaire pour assurer la viabilité de leur production agricole. Par ailleurs, la séparation de la vente et du conseil a prouvé, à l'usage, sa totale inefficacité ; c'est la raison pour laquelle je n'ai aucun mal à revenir sur l'une des recommandations que

remise à l'occasion de cette proposition de loi, nous a indiqué que cette séparation avait peu d'incidences sur les ventes. Elle peut en revanche freiner l'adoption des produits de biocontrôle et ainsi éloigner les agriculteurs des innovations. Il me semble que c'est un point important. En réalité, je pense comme vous que les agriculteurs ont besoin d'être accompagnés.

beaucoup d'autres secteurs pourraient être reconnus comme tels- je pense notamment à la santé ou à l'éducation. En outre, nous nous interrogeons sur la mise en oeuvre de ce dispositif et sur ses conséquences. Une fois de plus, l'absence d'une étude d'impact est préjudiciable sur de tels sujets. En effet, puisque, au-delà de deux refus, un demandeur d'emploi peut perdre ses droits à l'allocation chômage, adopter cet article revient à considérer qu'un demandeur d'emploi doit être mobilisable- quels que soient sa formation, ses aspirations ou son âge -pour aller travailler dans les champs. Pour les sénateurs de mon groupe, cet article 19, couplé aux articles 20 et 22, participe de la mise en place d'une approche clairement libérale du marché du travail, approche que nous ne soutenons pas sur le fond et qui, sur la forme, aurait nécessité un texte spécifique accompagné d'une réelle étude d'impact.

Assurer une orientation active des demandeurs d'emploi vers les secteurs prioritaires en tension identifiés par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

privée d'emploi à partir de son vécu et de son expérience professionnelle, pour mieux la réorienter ; non, on lui dira : « C'est là qu'il faut aller

aux parcours, aux aspirations et aux compétences du demandeur d'emploi. Mais l'article 19 ne remet nullement en cause cette nécessité ! Il a aussi été souligné qu'il convient de réfléchir à l'attractivité des conditions de travail dans les secteurs en tension, ainsi que d'accompagner les très petites entreprises pour la construction de fiches de poste. Une fois encore, l'article 19 ne remet nullement en cause cette nécessité. En revanche, il apparaît nécessaire- tel est bien l'objet de cet article -d'envoyer un signal et de permettre une orientation

voir les résultats de l'agence d'insertion du RSA que nous avons installée dans le département des Yvelines. On y assure un accompagnement des allocataires du RSA vers les secteurs en tension dans le département, vers les les entreprises qui acceptent de réintégrer ces travailleurs. Cela fonctionne extrêmement bien. Je trouve qu'il n'y a rien de choquant à accompagner des personnes privées d'emploi vers des secteurs d'activité qui recrutent. C'est pour ces raisons que l'avis de la commission sur ces amendements

dernière réforme de l'assurance chômage, les conditions d'accès à l'aide au retour à l'emploi ; l'attractivité de ces emplois a donc chuté. Il est illusoire de continuer de croire qu'il suffira de contraindre les demandeurs d'emploi à combler les emplois vacants, sans se demander pourquoi ceux-ci sont vacants.

Le scrutin est ouvert.

Par ailleurs, il faut également avoir à l'esprit que les métiers agricoles nécessitent des connaissances, des compétences et, aujourd'hui, le plus souvent, des formations particulières. En conséquence, cet article revient à considérer soit que le métier d'agriculteur ne nécessite pas de compétences ni de formation et, partant, que n'importe quel Français peut demain l'exercer- nous ne pensons pas que ce soit l'opinion des auteurs de cette proposition pour la plupart attachés au monde agricole et connaissent parfaitement ses problématiques -, soit que seuls les métiers les moins qualifiés et donc, bien souvent, les plus difficiles physiquement et les plus précaires, bien sûr, seront visés par cette expérimentation. C'est bien sûr sur ce second point que le bât blesse, et c'est pourquoi nous proposons la suppression de l'article 20.

présenter l'amendement n° 101. Cette proposition de mettre en place un cumul du RSA et d'un revenu d'activité dans un objectif d'insertion part d'un diagnostic complètement erroné. Les personnes éloignées de l'emploi le sont en raison de multiples facteurs : santé, mobilité, qualification, logement C'est plutôt sur l'accompagnement qu'il faut axer les politiques publiques, si l'on veut permettre ce retour à l'emploi. De plus, les problèmes d'appariement entre emplois vacants et demandeurs d'emploi sont avant tout dus à des problèmes d'attractivité des postes proposés- on l'a déjà dit -en termes de conditions de travail de salaires, problématiques majeures qui ne sont pas prises en compte par ce dispositif. Par ailleurs, celui-ci pourrait donner lieu à des effets d'aubaine complètement contre-productifs.

En bref, celui-ci alimentera la précarisation du travail en agriculture et ne renforcera pas son attractivité, bien au contraire. Il convient à l'évidence d'expérimenter d'autres voies, comme un revenu garanti décent, des mesures concrètes d'accompagnement à l'insertion des personnes éloignées de l'emploi

pour la faire converger plus nettement avec la proposition de loi de notre collègue Claude Malhuret qui a été adoptée dans cet hémicycle le 15 avril 2021,

57 % étaient considérés comme « difficiles » du fait du manque de main-d'oeuvre. Il y a donc là un vrai sujet sur lequel les articles 19 et 20

y fait l'objet d'une évaluation et les premiers résultats sont extrêmement encourageants. C'est pourquoi il convient d'inciter à la généralisation de ces expérimentations, qui visent à remettre le pied à l'étrier des bénéficiaires du RSA et- pourquoi pas ? -à susciter des vocations agricoles. Il y a aussi une vertu pédagogique dans le lien particulier d'un agriculteur avec les

Monsieur le ministre,

métiers parfois pénibles et dangereux. Surtout, le Président de la République a annoncé la plantation de 1 milliard d'arbres d'ici à 2030, ce qui nécessitera beaucoup de main-d'oeuvre en forêt pour préparer les terrains, procéder aux plantations et appliquer les protections nécessaires

». L'article L. 722-1 du même code précise que les « établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production

saisonniers, de la faiblesse des revenus agricoles et des conséquences économiques liées aux différentes crises- sanitaire, climatique et géopolitique -qui ont marqué le secteur ces deux dernières années. Alors que le Gouvernement a acté la prolongation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2025, cette proposition de loi le pérennise et étend le champ de ses bénéficiaires.

Rappelons que le dispositif TO-DE profite en premier lieu aux filières à haute intensité en main-d'oeuvre- arboriculture, maraîchage, viticulture, grandes cultures -au travers de contrats très concentrés dans le temps, pour un coût total de 561 millions d'euros en 2023- ce n'est pas rien !

Pour quel résultat ? Depuis 2010, le dispositif a-t-il réellement permis de lutter contre le travail illégal et le recours aux travailleurs détachés ou amélioré les performances économiques et sociales de l'agriculture française, notamment en termes de créations effectives d'emplois ?

travail, relatif à la minoration ou à la majoration des taux de contributions des employeurs applicables aux contrats courts, les entreprises agricoles et agroalimentaires dont l'activité est directement déterminée par le cycle naturel des récoltes. Nous souhaitons rappeler que la logique de ce dispositif dit de bonus-malus sur les contrats courts est d'encourager les entreprises à privilégier le recours à des emplois stables- CDI, CDD de longue durée ou contrats d'insertion. En conséquence, l'exemption des entreprises agricoles et agroalimentaires revient mécaniquement à encourager ces entreprises à recourir à des contrats précaires. Par ailleurs, même si les spécificités du secteur agricole en matière de besoin de main-d'oeuvre sont réelles, l'extension du champ d'application de cet article à l'ensemble des entreprises agricoles et agroalimentaires semble fortement disproportionnée. Nous proposons donc de supprimer cet article.

Les travailleurs saisonniers sont consubstantiels à l'ensemble de la production saisonnière, en particulier pour le maraîchage ou l'arboriculture. Il est évident que l'application du bonus-malus viendrait perturber et pénaliser

au changement de pratiques, puisqu'il est défini en tenant compte de la moyenne des pratiques du secteur. Ainsi, le taux de séparation de l'entreprise est comparé au taux de séparation médian de son secteur : l'effort demandé aux entreprises est donc particulièrement limité, alors que des solutions existent pour créer des emplois pérennes dans le secteur de l'agroalimentaire et faire face à la saisonnalité. Je pense notamment à la mise en place de groupements d'employeurs afin de limiter le recours aux contrats précaires.

Cet amendement vise à renforcer le présent article en revalorisant les augmentations proposées du crédit d'impôt permettant de financer le recours au service de remplacement. Actuellement, grâce à ce crédit d'impôt, les éleveurs et paysans contraints à une présence quotidienne sur la ferme peuvent bénéficier d'un financement égal à 50

Concernant le crédit d'impôt pour congé, l'amendement tend à fixer le taux de financement à 90 % pour la première semaine de congé, puis à 75 % pour la deuxième et troisième semaine. En effet, encore trop d'agriculteurs ne prennent aucun congé sur l'année, du fait de contraintes économiques : dans la version actuelle du crédit d'impôt, le reste à charge est trop important pour nombre d'agriculteurs, qui ne peuvent accéder au dispositif. Le mécanisme proposé leur permettrait de prendre une

alors que les agriculteurs souffrent trop souvent de conditions de travail difficiles et d'épuisement psychologique, avec les conséquences sur la santé et le risque d'accident que cela implique. Revaloriser fortement le crédit d'impôt permettrait de renforcer l'attractivité du métier d'agriculteur, alors que la France est confrontée à l'enjeu crucial du renouvellement des générations, et de créer des emplois durables dans les services de remplacement, acteurs essentiels pour la dynamique des territoires ruraux. Merci, la portée de l'article 23, qui tend à pérenniser et à augmenter le crédit d'impôt pour dépenses de remplacement applicable à certains exploitants agricoles. Il semble en effet indispensable de redonner de l'attractivité à la profession agricole du fait de l'enjeu crucial de renouvellement des générations et de l'installation des agriculteurs. l'accès au congé est capital, car il s'adresse notamment aux agriculteurs contraints à une présence quotidienne sur la ferme. Cet amendement tend donc à aller plus loin que le texte issu de la commission, en portant le taux des dépenses engagées au titre du remplacement de 66 % à 75

en portant le taux de 50 % à 66 % en cas de congé pour convenances personnelles et de 60 % à 70 % en cas de congé pour maladie. Par ailleurs, nous avons ajouté trois jours supplémentaires de congé pour formation

effet de favoriser la cession d'entreprises agricoles au bénéfice des jeunes agriculteurs, dans un contexte de décroissance du nombre d'agriculteurs. Il y va de la survie de la profession ! Quel

? ... La séance est levée.